J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la délégation sénatoriale à la prospective a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

Nous avons tous été indignés par ces saccages et les avons condamnés avec la plus grande fermeté. Les maires dont les bâtiments publics ont été vandalisés ont considéré qu’une minorité d’individus ne devait pas porter préjudice à l’ensemble de la population. entrepris au plus vite des travaux pour réparer et rouvrir le plus rapidement possible les écoles publiques, les centres sociaux ou même leurs mairies, qui ont été saccagées. Les assureurs disent désormais ne plus pouvoir prendre en charge ce type de contrat avec les collectivités territoriales et répondent de moins en moins aux appels d’offres. Quand certains décident finalement de le faire, ils proposent de nouveaux tarifs indécents. Les communes subissent une explosion de leurs cotisations ou de la franchise de leur assurance. Certaines ont même vu leur contrat résilié. C’est une très mauvaise nouvelle, une de plus pour les maires, qui doivent déjà faire face à bien d’autres difficultés financières. Élisabeth Borne, alors Première ministre, avait annoncé le 26 octobre qu’une enveloppe de 100 millions d’euros serait débloquée pour aider les villes à se reconstruire, et ce lorsque le reste à charge serait particulièrement élevé.

Le Sénat a aussi lancé une consultation en ligne des élus locaux afin de recueillir leurs témoignages. Après les émeutes de l’été dernier et la répétition des catastrophes naturelles, les communes sont très exposées et attendent des réponses fermes du Gouvernement.

Les deux ordonnances prévues par cette loi ont été adoptées en conseil des ministres dès le 13 septembre. Sur le plan financier, ensuite, une circulaire a été adressée dès le 7 juillet, c’est à dire au lendemain des événements, afin de préciser les modalités d’accompagnement des collectivités pour la réparation des dégâts. Le fonds dédié annoncé dans cette circulaire, qui doit venir compléter les remboursements octroyés par les assurances, a été abondé par des ouvertures de crédits en loi de finances de fin de gestion pour 2023 et a fait l’objet d’une seconde circulaire publiée le 20 décembre. Au total, 106 millions d’euros ont été rendus disponibles pour l’accompagnement des collectivités territoriales. Parallèlement, le travail a été engagé avec les collectivités et les assureurs afin d’évaluer les réparations à effectuer.

Au titre de l’année 2023, près de 20 millions d’euros ont d’ores et déjà été engagés au profit des collectivités qui soit n’étaient pas assurées, soit connaissaient déjà précisément le montant de leur indemnité d’assurance. Les collectivités qui n’ont pas encore reçu de subventions au 31 décembre sont celles qui sont assurées et qui ne connaissent pas pas encore le montant de leur indemnité d’assurance. L’État, à travers ce fonds exceptionnel, a en effet vocation à couvrir le reste à charge des collectivités après intervention des assurances. Afin de tenir les engagements pris

pour 35 kilomètres de lignes, 900 voyageurs par jour, 12 allers retours quotidiens, une desserte pour les salariés du Vimeu, des correspondances à Abbeville et la remise en service de la liaison entre Laon, dans l’Aisne, à l’est de la Picardie, et le littoral normand et picard. Si les promesses font saliver, l’addition est bien salée ! Le vent Le vent de jeunesse des mobilités va t il enfin souffler dans le nord de la France ? Je rappelle que nous sommes la première région éolienne de France. En effet, malgré la contestation des élus et des habitants, la région contribue en la matière aux objectifs fixés par le Gouvernement. il faut ajouter les deux réacteurs nucléaires EPR de nouvelle génération et la ligne à haute tension de transport, qui a un impact sur l’ouest du territoire, engagé dans cette transition écologique. Si je ne me trompe, c’est l’État qui a la responsabilité du financement des infrastructures. Le ping pong sans fin devient inquiétant, même si l’élan olympique est au goût du jour à la veille des jeux. Aidez les territoires ruraux ! La promesse est l’un des moyens de lutter contre ce qu’Hannah Arendt appelait « la chaotique incertitude de l’avenir », mais la promesse reste pour vous un îlot de sécurité.

et de la région Hauts de France. Elle fait partie des lignes couvertes par le protocole d’accord entre l’État et la région sur l’avenir des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire, signé le 18 mars 2022. Ce dernier prévoit que les investissements de régénération seront cofinancés par la région, à hauteur de 80 %, et par la sphère État, à hauteur de 20 %. Dans le cadre du contrat de plan État région 2015 2022, les études d’avant projet sommaire de réouverture de la ligne ont été réalisées. Depuis, la région Hauts de France a délibéré, le 23 novembre 2023, sur un projet de protocole d’accord concernant l’intégration du volet mobilité 2023 2027 au CPER 2021 2027 n’incluant pas le projet de réouverture de la ligne Abbeville Le Tréport. À ce stade, l’État n’a pas formalisé son accord sur ce protocole. Néanmoins, un accord pour la poursuite des études sur la restauration de la liaison a été conclu à la fin de 2023 entre l’État et la région. Ces études, qui seront à l’ordre du jour du prochain comité de pilotage prévu le 8 février, n’excluront aucun scénario de desserte. Cet accord traduit la continuité du soutien de l’État au développement de l’offre de transports la plus pertinente au service des usagers de la ligne Abbeville Le Tréport, sachant que c’est à la région, en tant qu’autorité organisatrice du transport ferroviaire régional, qu’il revient de définir cette offre. La parole

la Guyane, comme les autres territoires ultramarins, souffre d’un déficit grandissant de production agricole. Selon les dernières données disponibles, elle importe tous les ans les deux tiers de son alimentation. Pourtant, son agriculture se développe et le nombre d’exploitations augmente régulièrement, tout comme la surface utile agricole, mais cela reste insuffisant pour accompagner une forte croissance démographique. Les freins sont connus : difficulté d’accès au foncier ; coût de sa mise en valeur ; réglementation phytosanitaire européenne inadaptée ; aides européennes fléchées principalement vers les cultures d’exportation, dont la Guyane ne bénéficie pas. S’il est un domaine de la production agricole qui cumule les difficultés, c’est celui de l’élevage. La production locale couvre ainsi 29 % de la consommation locale pour ce qui est de la viande de bœuf, et à peine 1 % – oui

le cadre duquel sont testées depuis 2018 en Guyane des solutions permettant la coexistence entre l’élevage et la faune sauvage, ne donne pas satisfaction. Il est illusoire d’imaginer éradiquer complètement les attaques de félins. C’est pourquoi il faut instaurer rapidement un régime d’indemnisation des prédations dues aux félins de la forêt amazonienne et, pour cela, soumettre rapidement à l’Union européenne une demande de révision du régime cadre d’aides d’État.

porte ! La parole est à Mme la ministre. Monsieur le sénateur Patient, le Gouvernement est sensible aux difficultés rencontrées par les éleveurs de Guyane confrontés à la déprédation par les félins de la forêt amazonienne, en premier lieu le jaguar et le puma.

Ce régime constitue effectivement une aide d’État au sens du droit européen. Aujourd’hui, le jaguar et le puma sont des espèces qui ne sont pas protégées, mais qui, tout en étant en principe chassables, font l’objet d’un quota zéro. quota zéro. Un éventuel changement de statut de ces espèces, qui soulève, entre autres problèmes, des questions de droit international, est en cours d’examen. Je rappelle qu’elles sont toutes deux considérées comme quasi menacées dans la liste rouge des mammifères de Guyane établie en 2017. Dans l’attente, le ministère apporte depuis 2022 un soutien financier à l’association Hisa, pour, qui conseille et sensibilise les éleveurs aux attaques de félins.

dite loi SRU. Malgré ses contraintes budgétaires et ses obligations en matière de prévention des risques naturels, elle a pourtant manifesté un engagement concret en faveur de l’habitat public, notamment par la construction de logements pour gendarmes. Ces logements sont essentiels pour le bien être des forces de l’ordre et, par extension, pour la sécurité de la région. Alors pourquoi ne sont ils pas pris en compte dans l’évaluation des obligations de la commune au titre de la loi SRU ? Cet oubli ne reflète pas la réalité des efforts consentis ni l’esprit de solidarité et de renouvellement urbains que la loi est censée promouvoir. promouvoir. Cette commune et, au delà, toutes les communes de France concernées par ce problème, mérite une politique qui reconnaisse et valorise pleinement ses efforts, une politique, qui, au lieu de sanctionner, encourage et soutienne les initiatives locales contribuant à l’offre de logements publics. Face à cette situation, madame la ministre, ne conviendrait il pas d’adapter enfin les critères de l’article 55 de la loi SRU pour y intégrer les logements de fonction, comme ceux de la gendarmerie, et ainsi valoriser l’engagement des communes en matière d’habitat public ? La parole est public ? La parole est à Mme la Monsieur le sénateur Blanc, les dispositions de l’article 55 de la loi SRU visent à satisfaire les besoins en logement des ménages les plus modestes et à leur permettre de se loger dans la commune de leur choix, tout en favorisant la mixité sociale par la constitution d’un parc abordable, réparti de manière équilibrée sur le territoire. À ce jour, le décompte des logements sociaux pris en compte dans le dispositif SRU s’appuie principalement sur le conventionnement à qui garantit la pérennité des logements destinés à des ménages modestes, sous condition de ressources et avec des loyers plafonnés, dans un cadre réglementaire homogène et transparent. Sont également intégrés des logements du parc privé soumis à un régime spécifique garantissant leur finalité sociale, ainsi que certaines structures d’hébergement. À cet égard, les logements sociaux faisant l’objet d’un droit de réservation du ministère de l’intérieur sont bien comptabilisés dans l’inventaire d’une commune, au même titre que tous les logements conventionnés.

pour le calcul du taux de logements sociaux utilisé dans le dispositif SRU. Aussi, même lorsqu’ils ne font pas l’objet d’un conventionnement APL, ces logements ne viennent pas dégrader la part sociale du parc d’une commune. Enfin, il convient de rappeler que la décision d’un préfet de prononcer la carence d’une commune n’est jamais la conséquence automatique d’une simple lecture de l’évolution de l’inventaire des logements sociaux sur une période triennale. sur un diagnostic approfondi des services de l’État sur l’ensemble des actions mises en œuvre par les exécutifs locaux pour développer une offre de logements abordables sur leur territoire. l’occurrence, pour prononcer la carence de Robion, commune qui ne compte que 7,23 % de logements sociaux sur son territoire, la préfète du Vaucluse a considéré que les éléments avancés par l’exécutif local ne permettaient pas de justifier que seuls 30 % de son objectif aient été atteints au cours de la période 2020 2022. Je vous remercie

En effet, l’article R. 428 27 du même code n’est plus en conformité avec la nouvelle rédaction du texte issu de la loi du 2 février 2023, dite loi Cardoux, du nom de notre ancien collègue sénateur, qui en fut l’initiateur, et visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Au terme d’une procédure, la cour d’appel de Nîmes a relaxé quatre chasseurs qui étaient poursuivis, sur la foi d’un constat dressé par des agents de développement avoir participé à une battue de petits gibiers au mépris des règles de gestion édictées dans le schéma départemental de gestion cynégétique et dans le plan de gestion. a ainsi fait droit à la demande en nullité soulevée par les contrevenants en se fondant sur l’absence de compétence des agents verbalisateurs sur ce territoire, qui ne justifiait pas d’une convention avec ladite fédération. Cette situation bloque l’exercice des fonctions confiées aux agents de développement des fédérations départementales des chasseurs dans le cadre de la lutte contre le braconnage. Vous l’aurez compris, je souhaite savoir dans quel délai le Gouvernement envisage de présenter un projet de décret au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, en vue d’une entrée en vigueur lors de la prochaine campagne de chasse 2024 2025, qui débutera le 1 juillet 2024. La parole est à Mme la ministre.

notamment au regard des dispositions de la loi du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. ce texte a ainsi renforcé les compétences des agents de développement des fédérations départementales des chasseurs. Cet article de la loi n’appelle pas de texte d’application et la nouvelle rédaction de l’article L. 428 21 du code de l’environnement, postérieur à la loi « engrillagement », n’entre pas en contradiction avec l’article R. 428 27 du code de l’environnement. Aucune situation de blocage de l’action des agents de développement des fédérations départementales des chasseurs n’a été identifiée, la loi Engrillagement ayant au contraire étendu leurs prérogatives. Aussi, il n’est pas envisagé de procéder

La réforme des journaux télévisés de France 3 à la rentrée 2023, dictée avant tout par des considérations budgétaires, a été dénoncée par les journalistes et les personnels. Ils la jugent insatisfaisante d’un point de vue éditorial et épuisante pour les personnels. La charge de travail a été reportée sur les équipes régionales, la durée des éditions des journaux télévisés ayant été allongée du fait de la suppression des journaux nationaux, ce qui a provoqué les mouvements sociaux de la fin 2023. Le service public de proximité, cœur de métier des antennes régionales de France Télévisions, est aujourd’hui menacé par ces conditions de travail, alors même que les téléspectateurs ont longtemps plébiscité l’information locale et régionale, au plus près du terrain, à leur écoute, et qu’ils souhaitent la voir perdurer.

Il me semble donc nécessaire qu’un dialogue soit engagé entre les journalistes, les autres personnels et la direction de France Télévisions, afin d’identifier les pistes d’amélioration éditoriale et organisationnelle. Par ailleurs, cette démarche ne pourra se faire sans un état des lieux des moyens humains et financiers nécessaires pour assurer une information de qualité.

et met en valeur tous les événements culturels régionaux, répondant en cela à l’attente forte exprimée par les Français pour davantage de proximité dans les programmes et les sujets traités. C’est d’ailleurs pour cette raison que les Français soutiennent très largement le service public de l’audiovisuel. Le renforcement de l’offre de proximité de France Télévisions et de Radio France figurait parmi les priorités qui ont été définies pour le secteur audiovisuel public en 2018 et qui ont été formalisées dans un contrat d’objectifs et de moyens (COM) 2020 2022, prolongé par un avenant d’une durée d’un an. Cette dynamique a vocation à être amplifiée pour la prochaine génération en cours de négociation, mais elle s’est déjà traduite par plusieurs réalisations, parmi lesquelles le lancement par France Télévisions, au début du mois de septembre 2023, de « Ici 12/13 » et « Ici 19/20 ». Ces éditions d’informations, pilotées depuis les régions, mêlent informations nationales et informations locales. Si ce projet répond aux objectifs fixés par le Gouvernement,

conscients des vives tensions – vous les avez rappelées – qu’il a suscitées au sein des équipes de France 3. La direction de France Télévisions a pris des mesures pour les apaiser, notamment grâce à un protocole d’accord qu’elle a signé avec quatre organisations syndicales La direction du réseau est pleinement engagée pour améliorer les conditions de travail des personnels de France 3 et être à leur écoute. Une période de transition et d’adaptation aura lieu jusqu’au printemps, à l’issue de laquelle un bilan sera effectué. D’ores et déjà, je

pour 2021, qui est venue modifier le fait générateur de cette taxe pour les communes. En effet, avant 2022, cette taxe était exigible douze mois après l’obtention de l’autorisation d’urbanisme si la taxe due était

vingt quatre mois après. La loi de finances pour 2021 a acté le report de la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement à la date d’achèvement définitif des opérations, au sens de l’article 1406 du code général des impôts, mettant les communes dans une situation très délicate. Ainsi, depuis le 1 septembre 2022, le fait générateur de cette taxe est non plus la délivrance d’un permis de construire, mais la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux. Ces nouvelles modalités de perception posent plusieurs problèmes aux communes en matière de recouvrement et d’encaissement, notamment en raison du retard excessif de la déclaration d’achèvement des travaux par les contribuables, voire de son absence, ou encore du retard d’exécution des chantiers. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, j’avais déposé un amendement, largement adopté en première lecture, qui visait à revenir au système antérieur. Il n’a malheureusement pas été retenu dans le texte définitif. Ainsi, la détresse des communes provoquée par cette réforme injustifiée et pénalisante demeure, alors même qu’elles sont confrontées à d’importantes difficultés financières. Aussi, pour alléger les charges des maires, mais également pour éviter le non recouvrement d’une taxe primordiale dans l’établissement des budgets communaux,

Celui ci n’a pas remis en cause l’économie générale de la taxe d’aménagement et n’a modifié ni son fait générateur, qui reste fixé à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme, ni l’encaissement par la collectivité. Les modalités de transfert ont consisté à rapprocher le processus de liquidation de la taxe d’aménagement de celui des impôts fonciers, qui sont d’ores et déjà gérés par la DGFiP. C’est dans cette optique que la date d’exigibilité de la taxe a été décalée à la date d’achèvement des travaux, et ce afin de faciliter sa liquidation et de développer des synergies avec la gestion des impôts fonciers.

Tout d’abord, le report de l’exigibilité est décorrélé de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, puisque la réalisation définitive des opérations s’entend au sens fiscal de l’article 1406 du code général des impôts, dans lequel une construction est considérée comme achevée lorsque l’état d’avancement des travaux est tel qu’il permet une utilisation du local conforme à l’usage prévu, sans attendre les travaux de finition. Dès lors, une construction est considérée

En clair, les différentes mesures mises en place permettent de sauvegarder les recettes locales. Toutes les études qui ont été réalisées ont bien confirmé l’absence d’effets négatifs du décalage

relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables imposent à certains parcs de stationnement d’intégrer un dispositif d’ombrage par des ombrières comportant des dispositifs de production d’énergies renouvelables ou des dispositifs végétalisés. Ces obligations sont codifiées aux articles L. 171 4 du code de la construction et de l’habitation et L. 111 19 1 du code de l’urbanisme. Elles prennent effet à des délais différents en fonction du caractère nouveau ou existant de la construction, mais aussi du type de gestion et de la superficie concernée. Or, en pratique, certaines prescriptions couramment inscrites dans les règlements d’urbanisme peuvent se révéler incompatibles avec l’installation d’ombrières de ce type au droit des parcs de stationnement. Il en est ainsi des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives, des caractéristiques de toitures, ou encore de la limitation du coefficient d’emprise au sol. Je pourrais vous fournir des exemples précis. Les échéances fixées par la loi apparaissent malheureusement peu conciliables avec une procédure de révision des documents d’urbanisme ou de contestation d’un éventuel refus d’autorisation. Les pétitionnaires concernés sont aujourd’hui dans l’impasse. Beaucoup ont différé le dépôt de leur demande en attendant que soit réaffirmée la primauté de la loi sur les règlements d’urbanisme. Monsieur le ministre, comment comptez vous résoudre cette difficulté, que j’espère passagère ? La parole est à M. le ministre.

(PLU) peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits, ou selon la nature des activités qui peuvent y être exercées. Il peut également prévoir une interdiction de construire. Toutefois, les ombrières sont nécessairement rattachées à un parc de stationnement, qui est lui même soumis à ces règles. Dans la pratique, si celles ci permettent la construction du parc de stationnement, elles ne feront pas obstacle à l’implantation des ombrières.

à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Toutefois, si le COS est définitivement abandonné, d’autres règles comme l’emprise au sol des constructions, avec l’application d’un coefficient, ou encore des règles de gabarit, peuvent présenter un caractère contraignant qui, lui, peut limiter l’implantation ou les caractéristiques dimensionnelles des ombrières.

de l’article 40. Sans attendre les résultats de cette analyse, lancée en début d’année, je rappelle que les porteurs de projets qui envisagent de remplir leurs obligations sans attendre les échéances imposées par la loi peuvent d’ores et déjà demander à bénéficier des possibilités de dérogations aux règles des PLU ouvertes par l’article L. 152 5 alinéa 4.

Les mines de charbon, acteurs énergétiques historiques, doivent pouvoir contribuer à cette transition écologique, notamment par le développement du photovoltaïque ou encore de l’usage

précise sur un territoire de 1 100 hectares, en indiquant de manière claire qu’on ne peut pas à la fois se retrouver avec une friche et ne pas se demander comment elle peut concourir à l’atteinte de nos objectifs. Je

Merci, monsieur le ministre,

de cette problématique réelle sur le territoire, alors que les objectifs doivent être atteints au plus vite. Je vous remercie sincèrement de votre réponse,

mairie. Il semblerait que les secrétaires de mairie déjà en poste en tant que contractuels ne puissent pas tous bénéficier du nouveau dispositif prévu par cette loi. Un secrétaire de mairie comptant dix ans d’expérience dans différentes communes, mais dont le grade est adjoint administratif territorial principal de deuxième classe, ne peut pas être stagiairisé en vue d’une titularisation : selon la loi, une telle opération n’est possible que pour le seul grade d’adjoint administratif territorial. Un certain nombre de petites communes fonctionnent pourtant grâce à ces contractuels, qui jouent un rôle essentiel, à la fois auprès des habitants et des maires, dont ils sont souvent l’unique collaborateur. Le texte voté en décembre dernier est un premier pas, et il a suscité beaucoup d’attentes. Au regard de la faible attractivité de ce métier, je vous demande d’examiner cette situation précise et de rendre possible une stagiairisation, en prenant en compte, par exemple, le nombre d’années d’expérience, et ce quel que soit le grade. La parole

exclusivement aux fonctionnaires exerçant ou ayant vocation à exercer ces fonctions. Elle n’a pas créé de nouvelles procédures de titularisation des contractuels.

a donc souhaité renforcer la liberté laissée aux employeurs territoriaux de choisir entre un fonctionnaire et un contractuel, en fonction de leurs besoins. Pour autant, un secrétaire de mairie peut toujours, comme n’importe quel contractuel, intégrer la fonction publique territoriale en passant les concours,

SNCF. N’ayant reçu aucune réponse de Clément Beaune à ma précédente question écrite du 29 décembre 2022, je tente ma chance à l’oral ce matin. Rendez vous compte depuis quelques années, la SNCF interdit aux musiciens qui transportent des instruments encombrants d’accéder aux TGV. S’il semble que le problème ait été réglé pour les violoncellistes, on ne compte plus les contrebassistes, harpistes ou tubistes qui, dans le meilleur des cas, ont dû payer de lourdes amendes ou, dans le pire des cas, ont été tout simplement interdits d’accès au train. Pour des raisons qui semblent liées à des mesures de sécurité, le règlement actuel limite le transport aux instruments tenant dans un étui dont les dimensions Cette politique d’interdiction n’est pratiquée par aucune autre société de transport ferroviaire en Europe. Eu égard à la valeur des instruments et aux modalités du service de livraison de bagages, de remplacement est hors de propos. La solution simple et immédiate pour toutes les parties semble être, au vu de la faible population concernée, la mise en place d’un simple avis de tolérance. Monsieur le ministre, pouvez vous enfin trouver une solution de bon sens et obtenir de la SNCF qu’elle arrête de persécuter les saltimbanques, qu’ils soient harpistes, contrebassistes, ou bien encore batteurs percussionnistes, comme votre serviteur ? La parole est à M. le ministre. Monsieur le batteur Hugonet

vous avez indiqué que, compte tenu de la taille moyenne ou petite d’un certain nombre d’intercommunalités, un véhicule législatif serait trouvé en 2024 afin de satisfaire à deux impératifs. Le premier est de ne conserver aucun système de communes isolées. Le second est de faire preuve de souplesse et de trouver un système de coopération, tel que le syndicat mixte, sans obliger à transférer la compétence à l’intercommunalité.

Ils ont des questions simples et directes. Qu’entendez vous par « commune isolée » ? Ces assouplissements seront ils limités, par exemple aux territoires hyperruraux et de montagne ? Si oui, qu’appelez vous un territoire hyperrural ?

ce coût s’élevait à 69 millions d’euros en 2023. En 2024, il sera de 82 millions d’euros. Cette augmentation, insuffisamment justifiée par SNCF Réseau, a été validée par l’Autorité de régulation des transports (ART) en février 2023. C’est cette décision que sept régions de France, dont la région Nouvelle Aquitaine, ont décidé de contester devant le Conseil d’État.

Aujourd’hui, certaines questions méritent d’être soulevées, d’abord sur la transparence : qui décide quoi ? Les régions n’ont aucune visibilité sur les montants réinvestis, territoire par territoire, dans le réseau ferroviaire. Demanderez vous à SNCF Réseau

Quelles assurances seront données aux régions sur l’affectation des recettes issues des péages et perçues par SNCF Réseau ? Le choc d’offre de mobilité est percuté par le mur budgétaire…

C’est ainsi que, le 3 octobre 2021, la rivière La Beaume, qui traverse la commune ardéchoise de Vernon, a connu une crue sans précédent. Ce n’est que quatre heures après les fortes précipitations tombées sur les communes situées en amont que Vernon a été touchée.

Pourtant, si les prévisions avaient été fondées sur les quantités de pluie réellement tombées sur le haut du bassin versant, l’intensité et l’heure de la survenue de la crue auraient pu être annoncées avec précision au au moins deux heures à l’avance dans la commune de Vernon. Cela aurait conduit le maire à prendre des mesures adaptées afin de prévenir la catastrophe et d’en limiter les dégâts. Interrogés, les services de l’État ont répondu qu’ils ne disposaient pas des moyens techniques permettant de réaliser cette évaluation en temps réel et qu’il appartenait aux élus de consulter les intensités de précipitation en amont afin d’évaluer eux mêmes le risque encouru. Monsieur le ministre, avec les formidables progrès en matière de calcul et l’essor de l’intelligence artificielle, serait il possible de créer un dispositif d’alerte des crues fondées sur les précipitations tombant sur les bassins versants, ce dont les élus auront de plus en plus besoin ? La parole est à M. le ministre.

Ce qui sera bon pour ce territoire sera bon pour l’Anjou et ce qui est bon pour l’Anjou est bon pour la France.

L’effet pervers de cette mesure est clairement identifié : plus le parc de logements d’une commune est vieillissant, plus il est composé d’habitat social, plus la commune est pénalisée financièrement par ces exonérations. Il est incompréhensible de vouloir multiplier le nombre de rénovations et, dans le même temps, de priver financièrement les communes qui engagent ces programmes de rénovation. C’est le cas de la Loire,

Cette situation n’est plus tenable, particulièrement pour les communes les moins favorisées. Le dispositif d’exonération confirme, une fois de plus, le désengagement de l’État en matière de logement, au détriment des finances locales. Monsieur le ministre, l’année dernière, le Sénat a formulé une quinzaine de propositions pour rendre aux élus locaux leur pouvoir d’agir. Certaines sont un plaidoyer en faveur de l’autonomie financière des collectivités territoriales.

dans votre ancienne vie, à la métropole de Saint Étienne ou ailleurs, vous savez bien que la construction d’un logement neuf social entraîne une absence de taxe foncière pendant des années. Une telle mesure n’est aujourd’hui pas remise en cause,

les appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est supérieur à 1,5 tonne doivent être immatriculés. Depuis 2013, la réglementation encadrant l’immatriculation des remorques est devenue de plus en plus contraignante. Elle a cependant un effet sur une tradition rurale historique : celle des corsos, des fêtes des laboureurs, des fêtes des bouviers. Ces fêtes populaires coïncident bien souvent avec l’arrivée du printemps. Ces défilés de chars fleuris symbolisent depuis 1870 la transmission d’un véritable savoir faire entre générations, à tel point que la tradition des corsos est désormais inscrite au patrimoine culturel immatériel de la France. À l’origine, ces chars étaient tirés par des chevaux ou des bœufs. La pratique traverse les siècles grâce aux fêtes des bouviers, encore très présentes dans mon département de la Drôme.

nécessitera que les véhicules immatriculés figurent au fichier des véhicules assurés (FVA). La fédération des festivals, carnavals et fêtes Drôme Ardèche m’a alerté sur les difficultés financières liées à toutes ces contraintes, qui risquent d’être fatales à une tradition

Monsieur le ministre, pour que la tradition rurale et populaire des corsos puisse perdurer, la réglementation encadrant l’immatriculation et l’assurance des remorques agricoles peut elle être aménagée ? Des autorisations préfectorales pourront elles être délivrées en ce sens ? La parole est à M. le ministre. Monsieur le sénateur Monsieur le sénateur Buis, je vous réponds avec beaucoup d’humilité, car, à dire le vrai, en me levant ce matin, j’ignorais à peu près tout des réglementations concernant les remorques agricoles et de leurs conséquences éventuelles sur les défilés traditionnels et festifs. Voici l’état

Cette obligation s’impose aux véhicules ou appareils agricoles rattachés à une exploitation agricole mis en circulation après le 1 janvier 2013. 2013. Un arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers est venu préciser les modalités de réception de ces véhicules, notamment pour en garantir la sécurité. Conformément au code de la route, les propriétaires de véhicules soumis à immatriculation doivent en faire la demande avant la mise en circulation sur la voie publique. Un véhicule mis en service, mais ayant toujours circulé en milieu fermé, devra être immatriculé le jour où il circulera sur la voie publique. Toutefois, les véhicules ou appareils agricoles remorqués

Alors que la sinistralité augmente, des assureurs se retirent du marché, un marché pas toujours concurrentiel, ce qui entraîne un phénomène de monopole défavorable aux communes. Pourtant, le recours aux assurances est une nécessité en raison des activités multiples de nos communes : pour la flotte automobile, la garantie des biens, la lutte contre

Dans mon département des Ardennes, les exemples sont nombreux, tant dans les petites communes que dans les grandes agglomérations. Ardenne Métropole a constaté une augmentation de sa cotisation de 50 %, la commune de Bogny sur Meuse a subi une augmentation de 15 % pour l’assurance de sa flotte automobile. Nombreuses sont les communes à dénoncer ces comportements unilatéraux et soudains, qui les placent devant le fait accompli. Toutes nos communes rurales sont ainsi exposées à ces difficultés. Cela contredit le principe du mécanisme assurantiel qui est d’aider tout le monde face aux aléas et aux risques de la vie. Monsieur le ministre, sans assurances, la libre administration des collectivités locales est compromise. Qu’envisagez vous pour que nos communes puissent s’assurer dans des conditions sereines et non exorbitantes ? Comment les aider à faire face aux pratiques de certains assureurs, aux cotisations élevées ? Que comptez vous faire face aux résiliations anticipées qui sont une source de déséquilibre dans les relations entre les communes et leurs assureurs ?

Aux côtés des maires, elles doivent faire preuve de disponibilité, de rigueur et de polyvalence, entre autres qualités. En contrepartie de leurs responsabilités et de leurs tâches importantes, elles bénéficient d’un traitement et d’une évolution de carrière tout à fait insuffisants.

attaché à accompagner les maires de votre territoire et à quel point les binômes maire secrétaire de mairie sont absolument indissociables. La plupart du temps dans l’ombre, ces couples font en sorte de régler les problèmes de la vie quotidienne, accompagnent les détresses et les désarrois parfois intimes des familles de la commune, s’échinent à essayer de comprendre les règlements administratifs, montent les stratégies qui permettent de défendre un dossier à l’échelon intercommunal, par exemple un dossier de demande de subvention

Le législateur, parfaitement conscient de la nécessité de tenir compte des moyens financiers de chaque collectivité, a maintenu la liberté de recruter des secrétaires de mairie parmi les trois catégories hiérarchiques de la

Je pense aussi à la création d’une nouvelle voie de promotion interne pour faire en sorte que les secrétaires de mairie de catégorie B puissent exercer ce métier sur la base d’une formation qualifiante. Monsieur le sénateur, vous serez le premier à repérer les domaines dans lesquels il faut des ajustements d’ordre réglementaire ou législatif. Je me réjouis de toutes ces occasions qui seront autant de prétextes pour passer du temps avec vous. Bravo ! La parole est à M. Hervé Maurey, pour la

Il est par ailleurs situé à une heure de route des principaux hôpitaux de recours qui sont à Nantes, Rennes et Vannes. De plus, le diagnostic de santé de ce territoire est connu pour ses indicateurs très défavorables : surmortalité importante, part des patients en affection longue durée supérieure aux moyennes régionale et nationale. Un audit réalisé il y a plus de deux ans préconisait la construction d’un nouvel équipement plutôt qu’une réhabilitation qui ne permettrait pas de répondre aux besoins.

Ce projet revu à la baisse, avec moins de surfaces, moins de services et de lits, a été extrêmement mal reçu par les élus et les usagers, qui ont le sentiment de se voir proposer un projet d’hôpital au rabais. Après tant d’atermoiements et de mépris envers le travail collectif des élus du territoire, je souhaite savoir à quelle hauteur l’État compte s’engager pour un établissement qui n’a pas bénéficié d’investissements publics depuis une vingtaine d’années et qui ne pourra pas assurer un niveau d’autofinancement suffisant. La

Dès qu’on le cherche, on le trouve ! Ce métabolite est classé cancérogène probable. Aussi, madame la ministre, entendez vous prendre des mesures d’urgence sanitaire, mais aussi soutenir les collectivités confrontées à la nécessaire dépollution de l’eau ? En effet, il y a un réel risque de fracture territoriale de la qualité de l’eau,

L’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle Aquitaine estime que la situation « n’a jamais été aussi grave ». Il manque en moyenne 30 % de médecins dans les 15 services d’urgences de Gironde, ce qui entrave la continuité du service

À Sainte Foy la Grande, la situation est gravissime : on a compté, au cours des mois d’avril et mai 2023, plus de 17 jours de fermeture ! Les patients de ces hôpitaux sont redirigés vers le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à plus d’une heure de route. Ce CHU lui même est désormais contraint de réguler l’accès aux services d’urgence. L’été, du fait de l’augmentation de la fréquentation des sites touristiques en Gironde et des indisponibilités accrues de personnel, faute de moyens complémentaires, l’ARS envisage de déshabiller Pierre pour habiller Paul.

par la désertification médicale. Dans de nombreux territoires de notre pays comme de mon département de Saône et Loire, de très importantes difficultés persistent pour les Français qui sont à la recherche d’un médecin traitant. Je peux témoigner du désespoir qui étreint les patients et leurs familles lorsqu’un médecin prend sa retraite sans remplaçant et que 2 000 patients partent à la recherche d’un nouveau médecin traitant sur un territoire déjà particulièrement sous tension. Cette situation conduit par conséquent à une saturation, voire à une obstruction de l’hôpital public voisin. Certes, dans de telles situations, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) prévoit bien une neutralisation des pénalités de remboursement pour les patients dont le médecin part à la retraite ou ferme son cabinet. Mais les jeunes, les nouveaux arrivants sur le territoire, ou encore ceux de nos concitoyens qui n’ont jamais eu de médecin traitant

Pour toutes ces raisons, au regard de l’extrême tension du système médical dans notre pays et de l’égalité de traitement entre patients que nous devons à nos concitoyens, je vous demande, madame la ministre, si le Gouvernement compte affronter rapidement la problématique du parcours de soins coordonnés en désert médical, de manière à offrir aux patients qui ne disposent pas d’un médecin traitant

Faute de place au sein de structures publiques, de nombreuses familles se tournent vers des associations et des professionnels non conventionnés. Ces associations offrent une prise en charge pluridisciplinaire, grâce à des orthophonistes, des psychomotriciens, des éducateurs spécialisés et des psychologues.

Merci pour vos éléments de réponse, qui sont en effets importants, mais vous me parlez de l’école inclusive ; moi, je vous pose la question des structures non conventionnées accueillant des enfants qui ne vont pas tous à l’école. Il y a bien un plan Autisme,

En Guyane, les plaquettes nécessaires pour stabiliser son état de santé manquaient cruellement. Il faut dire que la Guyane est actuellement confrontée à une forte épidémie de dengue, qui rend plus complexe encore la gestion déjà difficile du stock de plaquettes.

transfusé aux Guyanais provient essentiellement des Antilles ou de la France hexagonale. Cette organisation pose plusieurs problèmes de santé publique. Se pose d’abord la question évidente de la disponibilité des stocks. En effet, la Guadeloupe n’est pas autosuffisante en matière de produits sanguins labiles. En outre, la France hexagonale et les Antilles se trouvent respectivement à huit et trois heures de vol.

multiplie les risques d’incompatibilité et de réactions transfusionnelles. Il y a deux ans, j’avais interpellé le Gouvernement sur cette même question. On m’avait opposé un rapport de Santé publique France. Or ce rapport ne ferme pas la porte à une reprise de la collecte du sang en Guyane ; il dit, tout au plus, qu’il y aura des contraintes.

d’être les sacrifiés ! Combien de Karen faudra t il, madame la ministre, avant que la France n’envisage sérieusement de reprendre la collecte de sang en Guyane ? Vous pouvez dès à présent, à tout le moins, autoriser le prélèvement des plaquettes, qui bénéficient d’un traitement rendant inactifs les virus. Ce sera un premier pas, en attendant que la recherche progresse

veux parler des difficultés liées à l’accueil des mineurs non accompagnés (MNA) et à leur entrée dans le dispositif spécifique qui leur est destiné, en amont de leur prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE). Les questions légitimement posées par les travailleurs sociaux restent globalement irrésolues à ce jour. Les cris d’alerte lancés par les départements sont laissés sans réponse. Pour faire bouger les choses, certaines collectivités, comme les départements du Territoire de Belfort, du Jura ou de la Vienne, adoptent des motions visant à limiter la prise en charge directe de ces mineurs étrangers. Deux difficultés majeures sont bien connues par les acteurs de terrain : la première est la phase d’évaluation des demandeurs, au cours de laquelle le placement en accueil provisoire d’urgence n’est pas toujours effectif ; la seconde réside dans la saturation des établissements d’accueil. Prenons l’exemple du Territoire de Belfort : on dénombre 61 places pour près de 90 mineurs non accompagnés. Madame la ministre, je ne vous apprends rien : cette tendance est très documentée, notamment par le ministère de la justice, qui, en septembre dernier, annonçait une augmentation du nombre d’arrivées de 30 % en 2022 par rapport à 2021. Pour toutes ces raisons, il me semble indispensable de procéder au transfert à l’État de la mise à l’abri des mineurs non accompagnés, comme le demande également l’association Départements de France. Madame la ministre, le Gouvernement compte t il prendre cette mesure, pour enfin soulager les départements au bord de l’asphyxie ? La

Madame la ministre, cette situation est courante en milieu rural et en montagne, où les distances parcourues et les temps de déplacement sont accrus. Elle se révèle particulièrement coûteuse pour l’assurance maladie et créée des ruptures de soins parmi ces patients, fragilisés par cette situation. Les cabinets libéraux contactés indiquent ainsi à regret que, dans un contexte inflationniste, le plafonnement de leurs indemnités kilométriques les empêche d’assurer une permanence de soins quotidienne dans des périmètres d’intervention plus éloignés. Au total, les dispositions prévues causent des inégalités d’accès aux soins qu’il apparaît nécessaire de prendre en considération de façon beaucoup moins technocratique, si possible dès la prescription de ces soins indispensables au bon rétablissement du patient, voire à son maintien à domicile. Supprimer des normes, réduire les délais, faciliter encore les embauches, augmenter tous les seuils de déclenchement d’obligation. C’est au fond la France du bon sens, plutôt que la France des tracas ». Madame la ministre, ces paroles sensées, prononcées par le Président de la République le 16 janvier dernier, résonnent tout particulièrement aux oreilles des habitants de la ruralité confrontés à ce « tracas » supplémentaire.

est aujourd’hui en péril et la mobilisation est générale, à l’échelon local, pour garantir la qualité et la continuité du service public de santé en Centre Bretagne. Il convient, une nouvelle fois, de souligner l’engagement sans faille et le dévouement incroyable des équipes de direction, des soignants et des praticiens hospitaliers, qui portent le CHCB à bout de bras. Madame la ministre, au regard de la gravité de la situation, quels moyens humains et financiers spécifiques l’État compte t il déployer dans les plus brefs délais pour permettre à chacun de naître, de bien vivre et de bien vieillir en Centre Bretagne ? La parole est à Mme

à l’établissement de diligenter une mission d’appui, pour analyser les difficultés rencontrées et surtout pour proposer des améliorations dans l’accès aux soins et l’organisation. Cette mission, dont

à cette situation, il faudrait qu’un décret d’application des articles L. 5125 6 et suivants du code de la santé publique permette aux agences régionales de santé – je sais qu’elles y sont favorables – de déterminer les territoires au sein desquels l’accès au médicament pour la population n’est pas assuré de manière satisfaisante. L’absence d’un tel décret m’apparaît d’autant plus absurde que, dans les deux villages que j’ai cités, il existe des infrastructures de santé et des cabinets médicaux. Ainsi, Saint Cyr sur Morin, situé dans un bassin de vie où habitent bien plus de 2 500 habitants, accueille un cabinet médical de sept professionnels de santé, qui réalisent plusieurs milliers de consultations.

Les traitements et les technologies qui existent sont coûteux et ont un effet négatif sur l’environnement. Tout est mis en œuvre pour assurer la distribution d’une eau potable conforme : c’est le cas en Charente Maritime, où des actions et des recherches proactives sont menées – mais à quel prix ?

Ainsi, l’État demande aux collectivités et aux sociétés délégataires productrices d’eau potable de trouver des solutions pour dépolluer, alors que pendant cinquante ans aucune recherche de toxicité n’a été entreprise. On sait par ailleurs qu’aucune mesure agronomique préventive ou d’amélioration des pratiques culturales

de l’environnement et du travail (Anses) a publié récemment les principaux résultats de la dernière campagne de mesures relatives aux polluants émergents dans l’eau potable. Le but de ces mesures est de détecter la présence de composés chimiques

ou vendus à d’autres entreprises. Or l’activité de location ou de promotion immobilière ne fait pas partie de l’objet social de l’AFD ; c’est donc un problème.

Alors que le développement des énergies renouvelables constitue un enjeu majeur pour notre souveraineté et que cet objectif est inscrit dans la loi, la petite hydroélectricité, énergie complètement décarbonée, héritage précieux déjà déployé sur l’ensemble du territoire national, dont la production représente l’équivalent de celle d’un réacteur nucléaire, a un rôle important à jouer dans la croissance de notre mix décarboné.

sur les 345 cours d’eau classés en très bon état, 337 l’ont été sans inventaire de terrain. En dépit du fait que cette faiblesse est bien identifiée, le dialogue se révèle encore parfois impossible avec certaines administrations. Ainsi, en Savoie, le projet de centrale hydroélectrique du Nant Rouge, qui est situé sur le territoire des communes de Crest Voland et de Notre Dame de Bellecombe, bien que lauréat de l’appel d’offres de la Commission de régulation

de terrain des cours d’eau versées aux dossiers des projets de petite hydroélectricité

l’assujettissement à la taxe d’habitation des maisons d’assistants maternels (MAM), mentionnées à l’article L. 424 1 du code de l’action sociale et des familles. Ces structures, au nombre de 4 500 dans notre pays, permettent à plusieurs assistants maternels

Dans une société où l’accueil des enfants en bas âge est un problème structurel qui pèse sur les dynamiques de la natalité, de telles structures gagneraient à être soutenues par la puissance publique. Or les MAM sont contraintes de s’acquitter de la taxe d’habitation comme s’il s’agissait d’une résidence secondaire et alors même que les assistantes maternelles exerçant à domicile en sont désormais exonérées. Ce prélèvement, qui grève une partie de leurs ressources, ne favorise pas leur développement et les place dans une situation injustifiée par rapport à d’autres structures, entreprises ou associations,

la crise avait mis en évidence la dépendance énergétique de la France, il me semblait indispensable de consolider à la fois nos filières de production énergétique et le développement durable, sans y sacrifier notre indépendance. Plutôt que de saisir cette occasion historique, le Gouvernement a, par arrêté ministériel du 26 avril 2023, rejeté la demande de concession formulée par la Française de l’énergie. Cette décision regrettable a été annulée par un jugement du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Strasbourg, qui a estimé que l’entreprise avait justifié de ses capacités techniques pour extraire du gaz de couche et de la qualité des programmes de travaux présentés pour démontrer que le gisement était exploitable. Cette victoire judiciaire a abouti au décret du 20 novembre dernier accordant la concession dite « Bleue Lorraine » jusqu’au 1 janvier 2040 et permettant le démarrage de l’exploitation d’un gisement équivalent à cinq années de consommation de gaz en France. Madame la ministre, si je me réjouis de cette décision, deux menaces planent encore

Madame la ministre, le méthane issu du gisement lorrain a une empreinte carbone vingt fois inférieure à celle du gaz de schiste fracturé importé des États Unis. Son exploitation permettrait la création de nombreux emplois, renforcerait notre souveraineté énergétique et traduirait notre engagement sur le plan écologique et environnemental. en cohérence avec sa politique économique et énergétique, le Gouvernement envisage t il de permettre pleinement à ce projet d’aboutir, en retirant l’appel qu’il a interjeté ? La parole est

de la souveraineté alimentaire. Madame la ministre, après l’expression de la colère de nos agriculteurs, voici celle de nos producteurs de miel. Hier, dans plusieurs départements, les apiculteurs se sont levés pour dénoncer la concurrence déloyale de produits importés qui déstabilisent le marché. La production de miel est en effet soumise à des contraintes conjoncturelles et structurelles qui inquiètent d’autant plus la profession qu’elles affectent un secteur dynamique comprenant plus de 70 000 apiculteurs. Sur le plan structurel, les organisations représentatives de la filière alertent sur l’importation de miel d’assemblage qui est parfois frelaté et dont la provenance

consommant 45 000 tonnes de miel par an. Ces difficultés s’ajoutent à une crise de la production, qui a été divisée par trois en vingt ans et qui est encore aggravée

dont nous ne pouvons que nous satisfaire. Mais cet accord, qui doit encore être adopté par les institutions européennes, ne sera effectif dans l’Union que dans deux ans. Alors, madame la ministre, pouvez vous nous dire ce que le Gouvernement compte mettre en œuvre à court et à moyen terme pour soutenir l’apiculture française ?

C’est la raison pour laquelle la France a soutenu, à l’échelon européen, le renforcement des exigences en matière d’étiquetage et de traçabilité du miel pour améliorer l’information du consommateur et lutter contre ce qui est une fraude.

fort impact sur la vie des communes concernées. Ce changement de statut pourrait résoudre les difficultés des éleveurs confrontés à la réglementation des chenils et il pourrait également permettre de les rassurer face à la mise en cause croissante de leur responsabilité lors d’incidents avec les randonneurs dans les estives et au sein même des villages. Madame la ministre, pouvez vous me confirmer que les chiens de protection, imposés dans le cadre du plan d’actions Ours brun, sont bel et bien, eux aussi, concernés par ce changement de statut ? Si oui,

Des travaux ont été engagés en ce sens de manière anticipée pour sécuriser les propriétaires et les éleveurs. Par exemple, les évolutions envisagées doivent permettre d’encadrer le régime de responsabilité pour éviter les recours abusifs et d’adapter la réglementation en matière d’installation classée pour la protection de l’environnement.

Je vous remercie, madame la ministre. Malheureusement, cette évolution n’épuisera pas le sujet de la prédation et du désespoir des éleveurs et des bergers qui voient, dans les Pyrénées, particulièrement chez moi en Ariège, leurs troupeaux décimés par les attaques d’ours.

plus de 760 000 patients, ce qui met en lumière les défis critiques de la gestion des services d’urgence : 90 % de ces services font face à des difficultés majeures et signalent des carences dans le personnel non médical. Le manque de médecins urgentistes a entraîné la fermeture des urgences de nuit, parfois plusieurs jours de suite, ou le week end dans mon département, le Vaucluse,

Il est impératif de prendre des mesures concrètes pour garantir la continuité des soins d’urgence et répondre aux besoins de la population. Le décès récent aux urgences d’Hyères du jeune Lucas, âgé de 25 ans, ignoré dans le couloir du service des urgences pendant des heures et découvert décédé au milieu des autres patients, en est l’exemple même. De tels drames ne devraient pas se produire dans notre pays, longtemps envié pour son avant gardisme en matière de soins. La vie de nos concitoyens dépend d’une réponse rapide et efficace. La désaffection de l’hôpital public, accentuée par des statuts moins attractifs et des rémunérations peu concurrentielles, complexifie la situation.

en ressources médicales. La mise en place de ce dispositif permettrait d’assurer la première urgence, souvent essentielle pour limiter les complications médicales qui sont parfois fatales – l’exemple

de garantir le soutien médical à nos forces armées et aux formations rattachées en tous lieux et en toutes circonstances ; il est le seul à pouvoir réaliser cette mission. Ce soutien se matérialise en opérations, où le SSA déploie une chaîne médicale opérationnelle pour la prise en charge de nos militaires quand ils sont blessés, de l’extrême avant jusqu’à leur évacuation vers l’Hexagone. Il se matérialise également sur le territoire national, où le SSA assure des missions de soins physiques et psychiques, d’aptitude médicale, d’expertise et de conseil aux commandements. Le SSA participe quotidiennement au système de santé grâce aux hôpitaux des armées : ceux ci accueillent environ 70 % de patients civils et contribuent pleinement à l’offre de soins, en lien étroit avec les ARS. Sous réserve de la priorité qui doit toujours être donnée à nos forces armées, le SSA peut être amené à mettre ses capacités

collège. Censé être un remède, ce « choc » suscite actuellement de très nombreux mécontentements, tant sur le recul pédagogique que constituent les groupes de niveau en français et en maths que sur les moyens attribués aux établissements pour le mettre en œuvre. Les dotations horaires dans mon département – mais c’est malheureusement le cas partout ailleurs en France – sont en effet très insuffisantes et la mise en place des groupes de niveau conduira à des classes surchargées surchargées dans des niveaux ou divisions ou dans d’autres disciplines que le français et les maths. Cela contraint aussi les collèges à puiser dans les ressources de dispositifs existants, alors que ceux ci sont importants pour l’apprentissage des élèves ou pour l’attractivité des établissements et qu’ils permettent de faire du sur mesure et de répondre à la réalité de chaque collège. chaque collège. À Fécamp ou à Saint Étienne du Rouvray par exemple, des collèges vont devoir supprimer des heures d’accompagnement personnalisé ou des dédoublements en langues ou en sciences. À Maromme, ce sont des classes qui devraient fermer. Quant au collège de Fauville en Caux, il devrait supprimer sa section de jeunes sapeurs pompiers. Je pourrais malheureusement citer bien d’autres exemples. Chaque année scolaire voit l’organisation des établissements bousculée ; les réformes se succèdent avant même que leurs résultats

Plus spécifiquement pour votre département, la Seine Maritime, dans le premier degré public, dans un contexte de baisse démographique – on a dénombré 7 509 élèves de moins entre 2017 et 2023 –, les taux d’encadrement se sont améliorés : le nombre d’élèves par classe est passé de plus de 23 à la rentrée 2017

à la rentrée 2024 ; malgré cette baisse, qui est significative, il ne devra restituer que 14 de ses emplois, garantissant justement les enseignements que vous avez décrits. Dans le second degré, les prévisions d’effectifs sont au contraire stables

le Gouvernement sur les difficultés rencontrées par les collectivités des outre mer dans le cadre des programmes gouvernementaux de revitalisation des territoires ruraux, tels que Petites Villes de demain et Villages d’avenir. d’avenir. J’ai été sensibilisé par le président de la communauté d’agglomération du pays Nord Martinique (CAP Nord), M. Bruno Nestor Azérot, sur la nécessité de renforcer les moyens humains, financiers et organisationnels inscrits dans les programmes gouvernementaux de revitalisation prévus pour ce territoire. M.

; enfin, créer un réseau d’échanges et de formation entre communes labellisées Petites Villes de demain et Villages d’avenir à l’échelle des Antilles et de la Guyane. Sur le fondement de ces éléments, je souhaite connaître les dispositions envisagées par le Gouvernement pour répondre au mieux aux attentes des élus des outre mer concernant les programmes nationaux de revitalisation des territoires ruraux. La parole

ultramarins entre les territoires, en compensant les obstacles liés à leur éloignement. Elle est fondée sur les principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République. La hausse brutale du prix des billets d’avion et du fret maritime depuis la fin de la crise sanitaire entraîne des difficultés majeures pour le déplacement des Ultramarins. Surtout, la politique de continuité territoriale est souvent envisagée sous le seul angle des liaisons directes entre les territoires d’outre mer et l’Hexagone.

ultramarins et les États voisins, non plus que, dans certains territoires, l’enclavement intérieur, en raison d’une desserte interîles peu diversifiée et onéreuse. En Guadeloupe, les îles du Sud, dont je suis originaire, sont reliées par bateau audit continent, Basse Terre et de Grande Terre, au moyen de traversées qui durent de trente minutes à une heure. Des aérodromes permettent aussi de relier ces îles, mais aucune compagnie ou presque n’exploite les liaisons entre la Guadeloupe « continentale » et les îles du Sud.

vers l’Hexagone. La politique de continuité territoriale a certes connu des progrès indéniables depuis ses débuts, voilà vingt ans. Néanmoins, elle reste très insuffisante pour répondre aux enjeux d’équité, d’égalité des chances et d’indivisibilité de la République.